La séance est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ont été publiées. J'informe également le Sénat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

L'article 1 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs a modifié les dispositions de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale pour permettre aux employeurs de moins de 20 salariés d'utiliser des offres de services simplifiées TESE et CEA. Ces offres étaient, jusqu'à la parution de l'ordonnance, réservées aux employeurs de moins de 9 salariés, à l'identique du régime applicable au dispositif « service emploi association ». Cette mesure doit permettre à toutes les têtes de réseaux associatives de continuer à bénéficier de ce service, malgré une augmentation de taille liée aux regroupements inhérents à l'adaptation à la nouvelle carte des régions, notamment. Elle doit aussi contribuer à soutenir le développement des groupements d'employeurs, désormais clairement reconnus comme facteurs de créations d'emplois. Ces groupements d'employeurs sont des associations susceptibles d'utiliser le dispositif « service emploi association pour faciliter leur gestion et leur développement. Le passage à 20 salariés me paraît indispensable pour leur permettre de continuer à y recourir après leur dépassement du plafond de 10 salariés. ministre, mes chers collègues, cette mesure doit permettre à cette offre d'être accessible à toutes les associations qui le souhaitent, malgré le nouveau décompte des effectifs. Ce dernier, intégrant de fait un nombre supplémentaire de salariés,

? Monsieur le rapporteur général,

La volonté actuelle du Gouvernement n'est pas de développer des dispositifs simplifiés concurrents les uns des autres pour une même population. Il est au contraire souhaitable, dans un objectif de simplification des démarches et de rationalisation des offres de service, mais aussi pour réaliser des économies au sein des organismes de la branche de recouvrement, de réduire la diversité de ces dispositifs et de les centraliser autour d'un système unique par population. Pour les associations, le Gouvernement souhaite travailler sur une convergence entre les deux dispositifs existants, pour aller vers une seule offre de service, alors que votre proposition tendrait plutôt à renforcer cette dualité de dispositifs. Dans l'attente, il est logique que l'offre Impact emploi, qui représente un accompagnement plus lourd que le chèque emploi associatif, soit réservée aux structures les plus petites. De plus, il ressort des chiffres à ma disposition qu'environ 15 000 associations employeuses utilisaient Impact emploi pour déclarer près de 36 000 salariés en 2016 et, ainsi, que la grande majorité de ces associations

les dysfonctionnements des dispositifs passés, même si quelques corrections avaient permis de diminuer le nombre de réclamations. Il reste à savoir si le nouveau schéma proposé permettra d'apaiser les inquiétudes, toujours vivaces, des indépendants comme des salariés. En défendant un amendement à l'article 4, j'ai pu dire combien notre groupe sera vigilant sur les conditions de mise en oeuvre de cette transformation et sur sa philosophie. En aucun cas, le changement opéré ne doit porter préjudice au régime général de la sécurité sociale, ni faire supporter des charges indues aux travailleurs salariés. Le premier enjeu est donc celui de la construction d'un système vraiment solidaire. Les auto-entrepreneurs, commerçants, artisans, sont bien conscients que leur intégration en deux ans au régime général posera, tôt ou tard, la question de l'harmonisation des cotisations et des prestations. Nous pensons, au sein du groupe CRCE, que la solidarité doit d'abord s'exercer entre les entrepreneurs eux-mêmes. C'est pourquoi nous regrettons vivement le refus du Gouvernement et de l'ensemble des autres groupes du Sénat de rétablir la contribution sociale de solidarité des entreprises, telle qu'elle a existé jusqu'en 2014 et dont le produit a malheureusement été réduit de 2 milliards d'euros Ce sont autant de recettes qui manquent à la sécurité sociale ! De plus, nous serons extrêmement vigilants sur les conditions de mise en oeuvre de cette réforme. Les salariés du RSI et des organismes associés attendent des garanties qu'ils n'ont pas obtenues jusqu'à présent. Or ce sont eux qui ont tenu à bout de bras un système défaillant ; ils espèrent une reconnaissance méritée de leurs efforts. En aucun cas, les salariés du RSI ne sauraient servir de « bouche-trous ». Leurs droits à une mobilité géographique, mais aussi fonctionnelle, réussie doivent être reconnus. Quels moyens, madame la ministre, monsieur le ministre, allez-vous mobiliser pour réussir cette transition, sachant que la carte des sites du RSI ne correspond en aucune façon à celles des centres d'assurance maladie ou des URSSAF ? Quels sont vos engagements en termes de compensations financières et de formation pour que chaque salarié soit respecté dans ses compétences actuelles et à venir ? Pouvez-vous vous engager à ce que les moyens de formation dégagés bénéficient à l'ensemble du personnel, et non à une cinquantaine de cadres, seulement, comme cela s'est malheureusement produit

sans réelle concertation et contre la volonté de ses administrateurs, des usagers, des syndicats, le Gouvernement a cédé à la pression médiatique et à la confusion entre poids des charges et méthodes de recouvrement.

lors, était-il nécessaire d'inclure dans le PLFSS un article de 30 pages et de plus de 400 alinéas, ne changeant rien sur le plan financier et ayant pour seule perspective une amélioration de fonctionnement déjà bien engagée depuis deux ans ?

L'usine à gaz initiée en 2008 à partir d'un logiciel obsolète, et qui était en voie de ralentissement, risque bien d'être réactivée. On peut s'interroger sur la constitutionnalité de ce texte : cavalier législatif peut-être ou convention de gestion déguisée ? Une saisine de la haute juridiction peut être envisagée. Oui, il fallait poursuivre une réforme en profondeur du RSI, mais en prenant le temps de la concertation pour aboutir dans un délai de deux ans à un projet de loi cohérent et accepté. Le réveil risque d'être douloureux. Nous prenons date.

des salariés, non que les responsables de l'époque aient voulu ainsi le limiter, mais, vous le savez, de nombreuses professions ont refusé de s'y insérer. Vint en 2006 le régime social des indépendants, qui concerne près de 4 millions de bénéficiaires et 2 millions de retraités, que le présent article vise à supprimer.

Jean-Luc Mélenchon -, « protection à deux vitesses »- Benoît Hamon -pour les autres, ou encore « catastrophe industrielle » pour la Cour des comptes- qui n'était pas candidate à la présidence de la République ... La suppression du RSI est donc réclamée d'une seule et même voix. Je ne peux que souscrire à la décision proposée. Les premiers concernés, les indépendants, rencontrent, en dépit des indéniables améliorations réalisées par le RSI, des difficultés persistantes. Celles-ci sont identifiées : erreurs dans les demandes de cotisations, recouvrements forcés, difficultés liées aux systèmes d'information, calculs de cotisations erronés, parfois cartes vitales non distribuées. Il est par ailleurs intéressant de constater que, chaque année, 400 000 nouveaux travailleurs indépendants sont affiliés au RSI, tandis qu'un nombre équivalent est radié et retourne vers le régime général. Les bénéficiaires du RSI évoluent au fur et à mesure du temps, et, parallèlement, leurs prestations se sont assimilées, par leur nature, à celles qui concernent les salariés. La suppression du RSI et l'adossement au régime général permettront, j'en suis persuadé, de mieux protéger les travailleurs indépendants en préservant notre modèle social, en garantissant les mêmes droits pour tous et en sauvegardant- c'est important -les spécificités liées à l'exercice de travailleur indépendant.

qui vont suivre devraient apporter des éclaircissements sur ces différents points. La parole est à M.

un véritable cauchemar aux travailleurs indépendants, aux commerçants, aux artisans et aux auto-entrepreneurs, qui ne représentent pas moins de 4,6 millions d'actifs et 2 millions de retraités. Le RSI, ou comment désarmer moralement, humainement, professionnellement 7 millions de professionnels, comment les dégoûter, les écoeurer de travailler, assommés qu'ils sont par des charges exorbitantes, équivalant à 50 % de leurs revenus pour certains entrepreneurs, ou, pis encore, par des cotisations supérieures à leur chiffre d'affaires pour certains ? Alors que dans le même temps, et dans un silence assourdissant, des centaines de milliers de personnes vivent de l'assistanat, des aides sociales, ... Oh ! ... devenues une véritable rente pour d'innombrables fraudeurs, et que des centaines de milliers d'étrangers- voire de clandestins -vivent aux crochets des finances de l'État Cette situation d'injustice est insupportable. Notre inquiétude est grande de voir de belles ambitions accoucher d'une souris. Certes, cet article supprime le RSI, mais il ne faudrait pas que celui-ci soit supplanté par un RSI. Car en réalité, il s'agit là d'un manque réel de simplification, alors que c'est le but de votre démarche et que c'est l'urgence absolue. Des inquiétudes se font jour, notamment au sujet des problèmes informatiques qui risquent de survenir. Elles portent aussi sur le fonctionnement du nouveau système, qui comprendra certes un guichet unique, mais trois caisses différentes. Un système éclaté très complexe, très coûteux, avec notamment un recouvrement des cotisations URSSAF alors que leur système informatique toujours en vigueur a prouvé ses défaillances. Mais plus qu'une fin du RSI, nous préconisons quant à nous d'offrir un véritable choix aux indépendants de s'affilier à un régime adapté à leur profession, avec des taux de cotisation raisonnables. Il faut leur offrir un bouclier social et la faculté de bénéficier, dès le 1 janvier 2018, de l'autodéclaration mensuelle ou trimestrielle. Voilà ce qu'attendent les travailleurs indépendants, car tous ne souhaitent pas être contraints de s'affilier à un régime général dont les taux de cotisation spécifiques semblent extrêmement précaires. Attention donc de ne pas nous précipiter. Les conséquences pourraient conduire les travailleurs indépendants à subir une situation plus compliquée et plus dommageable encore.

la protection sociale des indépendants, chargé de l'action sociale et de piloter le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire propre aux indépendants.

la désignation, par les instances régionales, d'un médiateur chargé d'accompagner les travailleurs indépendants et de les aider à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général. financement des actions de ses instances régionales avec des dotations annuelles attribuées par les branches maladie, vieillesse, complémentaire vieillesse et assurance invalidité-décès, le montant étant fixé par arrêté des ministres

qu'il est primordial de veiller au maintien des taux spécifiques qui étaient appliqués aux indépendants. Je me réjouis que le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants qui est créé reprenne le rôle social que les caisses régionales jouaient avec des dotations pour la prise en charge de cotisations pour les indépendants en difficulté. De plus, la version initiale se traduisait par une hausse des cotisations retraite pour les professions libérales. Un amendement

Durain. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la réforme précipitée du régime social des indépendants en 2008, bien que l'une des plus importantes réformes de structure et de simplification pour les usagers dans l'histoire de la sécurité sociale, s'est traduite par des dysfonctionnements graves.

des calculs de cotisations erronés liés à l'incompatibilité des systèmes d'information de l'URSSAF et du RSI, des difficultés rencontrées par les indépendants pour communiquer avec le RSI, une couverture santé jugée insuffisante. Les exemples sont nombreux. Ce constat est partagé par tous ; il a même été au coeur des programmes des différents candidats à l'élection présidentielle, ce point ayant également été rappelé. Compte tenu de l'ampleur des dysfonctionnements qui l'ont caractérisé au cours des dix dernières années, c'est une bonne chose que les candidats y aient prêté attention. Il importe désormais d'apporter sur le long terme la réponse que beaucoup attendent. Alors faut-il supprimer le RSI de la sorte ? Nous pensons en effet qu'une réforme d'ampleur du RSI s'impose, mais que l'ampleur d'une telle réforme justifie qu'elle ait lieu dans le cadre d'un projet de loi distinct d'une loi de financement de la sécurité sociale. Car nous ne sommes pas en train de discuter d'une variable d'ajustement budgétaire. Nous parlons d'un sujet majeur, qui mérite qu'on prenne du temps : du temps pour une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, du temps pour garantir l'opérationnalité des décisions à prendre. Ne nous leurrons pas : une telle suppression risque d'entraîner des dysfonctionnements techniques tels que ceux qu'ont connus les affiliés au RSI lors de sa création, dysfonctionnements souvent liés à une incompatibilité des systèmes d'information, et qui justifient aujourd'hui en partie la suppression du régime. Donner du temps à la suppression du RSI, c'est prendre les mesures nécessaires et mettre les moyens suffisants pour améliorer les systèmes d'information, notamment s'agissant du recouvrement des cotisations. Pour les assurés comme pour les personnels des caisses de sécurité sociale, il est indispensable que toutes les garanties soient réunies. Madame la ministre, mes chers collègues, nous estimons que cet article 11 est un cavalier législatif. En effet, l'essentiel, les dispositions qui figurent dans cet article portent non pas sur les règles relatives à la maîtrise des dépenses sociales et de santé, qui sont pourtant l'objet des lois de financement de la sécurité sociale, mais sur l'organisation, la gouvernance, la représentation des assurés, les règles d'affiliation, de prestation et de cotisation d'un nouveau système de portée générale.

Elle permet à la fois de sécuriser le transfert des assurés sans pour autant ouvrir une période trop longue qui insécuriserait notamment les personnels. Ceux-ci souhaitent, et on les

et que cette réforme se fasse rapidement pour qu'ils puissent avoir une affectation au plus près de chez eux, ce qui leur est garanti. Notre commission a adopté la semaine dernière une série d'amendements visant à préciser le dispositif et à permettre au Gouvernement de s'expliquer au cours de cette séance, en particulier sur le pilotage de la réforme.

également un engagement du Président de la République pendant la campagne. Nous sommes évidemment très vigilants afin de réussir cette réforme, et nous avons donc tenu compte de l'expérience du passé. Nous nous donnons le temps qu'il faut pour la réussir, avec une organisation dédiée. La première étape, vous le savez, c'est une période transitoire de deux ans qui permet de faire évoluer les organisations de travail, de négocier la transition avec les représentants du personnel- j'y reviendrai dans un instant plus spécifiquement à M. Watrin. Pour la reprise des missions des organismes conventionnés, la bascule se fera dans le courant de l'année 2020. Nous avons donc une période de deux ans pour aboutir au schéma cible. Pour les systèmes d'information, nous ne fixons pas de date butoir : l'évolution se fera progressivement au fur et à mesure de la maturité des projets. Nous nous donnons également des outils pour réussir cette réforme. Depuis le mois de juillet, une mission IGAS-IGF de préparation et de pilotage de la réforme, présidée par Dominique Giorgi, que vous avez auditionné, élabore le projet stratégique d'organisation prévu par la loi. Pendant la période de transition, le pilotage opérationnel sera assuré par les organismes du régime général, avec un comité de surveillance chargé de valider chaque grande étape du changement. Pour les systèmes d'information, nous avons mis en place un groupement d'intérêt économique formé par les différents organismes du régime général pour maintenir et faire évoluer en commun les applicatifs du RSI.

outre, concernant les personnels du RSI, vous avez raison, monsieur Watrin, ils n'ont pas à faire les frais de cette réforme. Ils ont fait des efforts considérables pour être devant les guichets au moment où le service dysfonctionnait. Nous sommes donc attachés à ce que cette réforme soit conduite de façon exemplaire pour eux. Nous avons pris l'engagement, évidemment, qu'il n'y aura aucun licenciement, aucune mobilité géographique contrainte. Nous avons donc prévu une période de transition de deux ans pour faire évoluer les organisations de travail et les contrats de travail. Pendant cette période, nous négocierons l'intégration des personnels dans la convention collective du régime général. Le projet de loi prévoit que les négociations seront engagées avant le 31 mars 2018. Il est prévu de négocier d'abord un accord de méthode, puis un accord d'accompagnement au changement, et enfin un accord de transition pour passer des conventions collectives du RSI aux conventions de l'Union C'est d'ailleurs l'accord d'accompagnement qui prévoira notamment les formations pour les personnels. Nous accordons donc au processus une très grande attention. Nous avons pris plusieurs fois ces engagements à la fois devant la représentation nationale et devant les représentants des salariés du RSI et des organismes conventionnés.

au cours de ces dernières années et lors de la campagne électorale, il a été abondamment dit qu'il représentait une difficulté majeure pour les indépendants, suscitant chez eux non seulement la colère, mais parfois même le découragement.

de simplification et de garanties pour les travailleurs indépendants. Non seulement c'est un engagement du Président, mais c'est aussi une demande persistante des indépendants, qui nous ont tous demandé au cours de ces derniers mois

L'enjeu pour le régime général, c'est d'accueillir les travailleurs indépendants en tenant compte de leur spécificité, qui se manifeste dans trois domaines : le recouvrement, l'action sanitaire et sociale et l'assurance vieillesse complémentaire, dont la gestion va à l'avenir à l'avenir incomber à la CARSAT. La forme que prendra cet accueil est à définir et peut-être, madame la ministre, pouvez-vous nous en dire plus à ce stade sur l'avancée des travaux. Ce qui me paraît essentiel, c'est de bien conserver une capacité d'accueil dédiée aux travailleurs indépendants au niveau des URSSAF pour le recouvrement et de la CNAV pour l'assurance vieillesse, car cette dernière aura à gérer l'assurance de base et la complémentaire des travailleurs indépendants. Au niveau de l'assurance maladie, il n'y a pas de changement, les prestations étant strictement identiques ; un service d'accueil dédié ne me paraît pas essentiel. L'objet de cet amendement est de préciser que le schéma stratégique d'organisation permettra la mise en place de cet accueil de répondre ainsi à l'inquiétude des travailleurs indépendants.

est ainsi libellé : La parole est à M. Stéphane Ravier. Cet amendement vise à offrir aux indépendants la possibilité de continuer à bénéficier d'un régime de protection sociale spécifique jusqu'au 31 décembre 2020, soit trois ans à compter de l'entrée en vigueur du texte. Ce délai permettra de préparer une alternative pérenne au régime général, de bâtir un nouveau régime social des indépendants qui leur garantira une couverture de santé et de retraite suffisante à des taux de cotisation adaptés. Comme pour la protection sociale des salariés, nous devons aborder la question du financement de la protection sociale des indépendants. La suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des sociétés pose la question d'un mécanisme de compensation qui prélèverait sur une partie des dividendes des grandes entreprises une contribution pour les artisans et les commerçants. Les travailleurs indépendants ont une culture propre qu'il faut respecter. Or les dispositions de cet article ne tiennent pas compte de leurs spécificités. Il faut se donner du temps pour construire une réforme ambitieuse et plus équilibrée qui conservera la liberté dont ont besoin nos petits petits commerçants, nos artisans et nos auto-entrepreneurs, tout en renforçant leur protection mise à mal par un modèle économique ultralibéral et hypermondialisé. Quel est l'avis de la commission ? Monsieur Ravier, si j'ai

monsieur le ministre,

est l'une des spécificités très fortes du RSI, est dotée d'un fonds de 115 millions d'euros par an et se structure autour de plusieurs axes l'aide à la complémentaire santé, l'aide aux cotisants en difficulté et l'aide au maintien à domicile. La mission sénatoriale d'évaluation et de contrôle sur le RSI, pilotée par Jean-Noël Cardoux et Jean-Pierre Godefroy, avait constaté l'attachement très fort des élus du RSI à ce dispositif. Aussi, madame la ministre, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les garanties offertes par le présent texte pour rassurer les travailleurs indépendants quant à l'avenir de leur action sociale et leurs capacités à conserver leur rôle de pilote, par l'entremise de leurs représentants ?

de l'action sanitaire et sociale. Il s'agit donc bien d'une compétence exercée en propre par ce conseil, et nous sommes favorables à votre amendement rédactionnel.

: La parole est à Mme la ministre. La suppression du RSI et l'affiliation des travailleurs indépendants au régime général conduit à la suppression des recettes propres de ce régime. Toutefois, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants supportera des dépenses de gestion administrative et continuera d'attribuer des aides et des prestations d'action sociale versées par les organismes du régime général. Le présent amendement précise les modalités de fixation des dotations et leur imputation dans les comptes du régime général, qui en assurera le versement.

allons lui rappeler ce que disait, il y a quelque temps, celui qui est devenu ministre de l'économie. Le présent amendement vise à créer un bouclier social pour les travailleurs indépendants. Il a été question de réduire les cotisations pour les travailleurs salariés, notamment pour ceux dont le revenu est au niveau du SMIC. Parlons à présent de ces travailleurs indépendants, qui sont appelés à cotiser alors qu'ils se retrouvent avec des revenus inférieurs au revenu de solidarité active, le RSA, c'est-à-dire l'apport de ceux dont la trésorerie est la plus fragile tentez d'aider ainsi des pépites de savoir-faire qui disparaissent, faute de soutien de l'État ! Rappelons que cette proposition avait été avancée, en son temps, par l'ancien député et actuel ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire. En septembre 2015, celui-ci déclarait- voyez, monsieur le ministre, à quel point mes références sont sérieuses Il faut créer un bouclier social pour que les indépendants ne se retrouvent pas avec un niveau de revenus inférieur au RSA à cause de cotisations excessives. » Par ailleurs, ce bouclier agirait comme un plafond, au-delà duquel les indépendants ne seraient plus appelés à cotiser davantage, et garantirait un revenu préservé pour les entrepreneurs. Il s'agit d'une mesure de bon sens pour aider nos travailleurs indépendants les plus fragiles. M. Le Maire I avait raison. Nul doute qu'avec M. Le Maire II, devenu ministre, vous vous accorderez sur cette ligne, afin d'envoyer un signal à beaucoup de nos concitoyens qui sont souvent à deux doigts de mettre la clef sous la porte de la commission, monsieur le rapporteur général, une telle exonération serait-elle permise ? Quelles seraient ses conséquences sur l'équilibre financier du régime ? De plus, ce dispositif rompt avec le principe de lien entre la cotisation et la prestation. Actuellement, 30 % des travailleurs indépendants sont déjà assujettis au paiement de la cotisation minimale. depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, un mécanisme de dégressivité a été introduit lorsque le revenu du travailleur indépendant est négatif ou nul.

Regroupant plus de 350 professions libérales différentes, la CIPAV gère près de 600 000 actifs cotisants, dont 320 000 exercent sous le statut de micro-entrepreneur, et verse les retraites de 100 000 affiliés. Les alinéas 209 à 218 de l'article 11 transfèrent au régime général environ 500 000 professionnels libéraux actuellement affiliés à la CIPAV, soit 90 % de ses ressortissants. Madame la ministre, la CIPAV a fait ses comptes. Ce transfert va conduire à une augmentation de 50 % des cotisations au titre du régime de retraite. Certes, des dispositions ont été adoptées par l'Assemblée nationale pour réduire durablement le taux de cotisation au titre du régime complémentaire. Mais, précisément, elles ne concernent que le régime complémentaire et non le régime de base. De plus, elles n'entrent pas dans le champ d'application d'une loi de financement de la sécurité sociale. En outre, ce taux réduit de cotisation, dérogatoire au droit commun, n'a fait l'objet d'aucun avis du régime complémentaire des indépendants et conduira à une réduction proportionnelle des droits à retraite complémentaire des professionnels libéraux qui demanderont à en bénéficier. En dernier lieu, ce transfert présente des risques importants. aux risques juridiques. Selon nous, cette mesure ne tire pas toutes les conséquences de la censure partielle, prononcée par le Conseil constitutionnel, de l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ces dispositions prévoyaient déjà le transfert d'un certain nombre d'affiliés de la CIPAV, mais, à l'époque, vers le RSI. Ensuite, je pense aux risques en termes de gestion

l'opération de transfert porte sur des enjeux financiers importants, de plus de 10 milliards d'euros. Pour autant, le texte est muet sur les conditions dans lesquelles vont être transférés les engagements de retraite des professions qui sont appelées à rejoindre le régime général. Enfin, le passage de 600 000 à 60 000 affiliés suscite, vous l'imaginez, l'inquiétude des 330 salariés de la CIPAV quant au maintien de leur emploi. Cet amendement tend donc à supprimer les alinéas 209 à 218 et, en conséquence, les mesures d'application correspondantes, qui figurent de l'alinéa 286 à l'alinéa 397. Le but est d'obtenir la suspension de la mesure aux fins d'un examen plus approfondi des contours, du contenu et du calendrier de la protection sociale des professions libérales.

texte, la semaine dernière, notre commission a adopté, par deux fois, le principe d'une limitation du périmètre d'activité de la CIPAV.

constitutionnel, en fixant dans la loi les professions qui demeureront affiliées à la CIPAV. Certes, il s'agit d'un dossier très sensible. La caisse a été, à deux reprises, sévèrement critiquée par la Cour des comptes, malgré le début d'amélioration constaté pour la qualité du service. La mission conduite par Philippe Georges a reconnu la difficulté à proposer une définition simple des professions libérales non réglementées. Le cantonnement du périmètre de la CIPAV devrait permettre de simplifier l'affiliation de certaines professions, pour lesquelles la limite est floue entre activité libérale et activité commerçante : il en est ainsi, par exemple, pour les prestations de services en informatique.

il peut percevoir des droits aux prestations en espèces maladie-maternité dans le nouveau régime qui sont calculés sur la base des périodes d'affiliation de son précédent régime. Ces prestations sont alors servies par le nouveau régime.

en espèces ne sont pas remplies, il demeure rattaché pendant un an à son précédent régime, auprès duquel il peut bénéficier des prestations en espèces. En l'état, cette nouvelle disposition pourrait entraîner des difficultés de gestion pour les régimes et avoir des conséquences sur les indemnisations des assurés. C'est dans cette perspective de la réforme du régime social des indépendants, le RSI, que le présent amendement vise à réintroduire les règles actuelles de coordination inter-régimes, lesquelles ont prouvé leur efficacité et sont plus adaptées, afin qu'elles continuent à s'appliquer.

la ministre pourra sans doute nous éclairer davantage quant aux limites de cet amendement, pour lequel la commission a décidé de suivre l'avis du Gouvernement.

En effet, en conséquence de l'adossement du RSI au régime général, il a été décidé de faire entrer, dans les conseils et conseils d'administration des caisses locales, un représentant désigné par les instances régionales du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La composition des conseils et conseils d'administration de ces organismes

présent amendement prévoit de toiletter les dispositions de l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 relatives aux transferts financiers entre régimes découlant des transferts de population organisés entre la CIPAV et le RSI.

rapporteur général. Cet amendement vise à renforcer le pilotage politique de la réforme par l'intermédiaire du comité de surveillance. Il permet, tout d'abord, d'instituer ce comité auprès des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget pour qu'ils supervisent directement le pilotage de la réforme.

doivent pouvoir être tranchés par les ministres, sans laisser la situation se dégrader comme cela a été malheureusement le cas en 2008 lors de la création de l'interlocuteur social unique- ISU -et de la méfiance mutuelle entre le RSI et les URSSAF.

la date d'extinction serait postérieure à celle de la fin de la période de transition, de façon à garantir que l'actuel système d'information du RSI ne soit débranché que lorsque le nouveau système est parfaitement opérationnel.

pouvez-vous nous en dire plus sur cette question fondamentale du système d'information ? On le sait, l'insuffisance du logiciel SNV2 avait été pointée pour expliquer l'échec de l'ISU. logiciel n'était toutefois pas le seul responsable, puisque la mauvaise qualité des bases de données du RSI au moment de leur transfert aux URSSAF a également eu des conséquences. Le travail de reprise de ces bases de données depuis dix ans permet d'être plus confiant dans le fonctionnement futur

par la mission d'accompagnement IGAS-IGF que nous avions mise en place en juillet. L'objectif est bien entendu de sécuriser le fonctionnement des systèmes d'information et de ne les faire évoluer que progressivement, au fur et à mesure que la bascule sur de nouveaux outils sera possible et validée. À cette fin, comme je le disais il y a quelques instants, les branches du régime général sont en train de constituer un groupement d'intérêt économique- GIE -, dont l'objectif sera d'assurer la maintenance des systèmes d'information du RSI tant que les évolutions nécessaires des applicatifs du régime général n'auront pas été réalisées. modernisation de l'action publique- le SGMAP -, est en cours pour identifier le schéma informatique cible à moyen terme. Les évolutions les plus importantes concernent la branche maladie. C'est pourquoi le transfert des organismes conventionnés vers les caisses primaires Sur la question du recouvrement et du logiciel SNV2 que vous avez mentionné, il n'est pas prévu de faire évoluer à court terme le système d'information de l'ACOSS, l'organisation du recouvrement s'étant améliorée et stabilisée au cours des dernières années avec une organisation spécifique.

Mme la ministre. Le présent amendement vise à simplifier le dispositif juridique lié à l'accomplissement des missions au bénéfice des travailleurs indépendants et à faciliter l'exercice des responsabilités confiées aux caisses déléguées, sans qu'il soit nécessaire de devoir recourir à une multiplication de délégations entre l'ensemble des organismes qui serait source d'insécurité juridique.

en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents aux organisations candidates à la désignation des membres des instances nationale et régionales puisse être établie en application de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, il convient de prévoir des mesures transitoires. Celles-ci, retenues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, risquent de conduire à ce que de trop nombreuses organisations puissent, pendant la période transitoire, siéger au sein de l'assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

C'est la raison pour laquelle, sans nécessairement aller jusqu'à demander la prolongation des mandataires actuels, il faut prévoir des modalités de désignation assurant une bonne maîtrise des thèmes qui seront abordés par les membres de ces instances. Tel est l'objet de cet amendement.

qui, combinées avec les nouvelles règles de désignation fixées dans le code, sont difficilement intelligibles. De plus, nous n'avons pas, à ce stade, une vision claire sur la projection des rapports de force dans les futures instances du CPSTI. Dans le champ des négociations nationales et interprofessionnelles, la fixation dans le code du travail du seuil minimal d'audience- 8 % des entreprises adhérentes à des organisations représentatives ou 8 % des salariés de ces mêmes entreprises -avait fait l'objet de concertations avec les partenaires sociaux. sociaux. Pour les travailleurs indépendants, une consultation spécifique sur la question de la représentativité n'a pas eu lieu. Dès lors, en renvoyant à un décret la fixation des règles de la mesure de l'audience et de la répartition des sièges

Je demande donc l'avis du Gouvernement, tout en émettant plutôt un avis défavorable pour ne pas perturber l'économie générale du dispositif qui me paraît toutefois insuffisant.

Il est prévu de reprendre, de manière quasi identique, les mécanismes en vigueur en droit du travail pour la mesure de la représentativité des entreprises. Ces mécanismes sont, par ailleurs, proches de ceux qui sont utilisés pour établir la représentativité des organisations participant aux négociations des conventions des diverses professions médicales. La loi prévoit bien qu'il y aura un seuil minimal d'effectifs pour établir la représentativité. Compte tenu du partage habituel entre la loi et le règlement dans le domaine de la sécurité sociale, la valeur de ce seuil sera fixée par décret. Le Gouvernement envisage bien de reprendre un seuil de 8 %, qui sera exprimé de manière similaire à celle qui est retenue en droit du travail pour établir la représentativité des organisations d'employeurs. Pour le reste, le décret reprendra les dispositions existantes en matière de droit du travail, afin de préciser notamment comment est traitée la situation des fédérations qui regroupent plusieurs organisations de base, les modalités de dépôt des dossiers, les justificatifs à produire- notamment dans quel cas sont requises des attestations de commissaires aux comptes -ou l'organisation des contrôles par l'administration des éléments déclarés.

vous indique que les conditions de désignation des représentants des travailleurs indépendants sont en cours d'élaboration. Ils ont fait l'objet de très nombreux échanges avec les différentes organisations. Le projet de loi prévoit que les membres du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales soient désignés sur la base d'une mesure de l'audience, prenant en compte le nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents. Un amendement adopté par l'Assemblée nationale a simplifié l'organisation de cette mesure d'audience, qui aura lieu courant 2018. Ce mode de désignation garantira la bonne représentativité des membres du conseil et de ses instances, ce qui est essentiel, et permettra une prise en compte adéquate au sein des instances de gouvernance des organismes de sécurité sociale des spécificités des travailleurs indépendants. Il ne nous paraît donc pas justifié de remplacer cette proposition par un autre mode d'organisation, qui nous semble plus coûteux et plus complexe.

Monsieur le sénateur, le terme de circonscription qui est utilisé dans l'article renvoie au périmètre géographique de compétence des organismes du régime général, auxquels vont être transférées les missions du RSI. La disposition figurant dans le projet de loi vise bien à garantir aux salariés du RSI qu'ils seront affectés dans l'organisme le plus proche de leur lieu de travail. L'écriture actuelle du texte répond donc à la préoccupation que vous exprimez et que nous partageons. C'est pourquoi

général. Avec cet amendement, nous abordons la question du transfert des personnels du RSI. Si notre commission n'a pas souhaité proposer un allongement de la période de transition, qui aurait pu laisser plus de temps aux organismes du RSI et du régime général pour mener à bien cette réforme, c'est en raison du risque d'évaporation des compétences, pour reprendre une expression entendue lors de l'audition des responsables du RSI. Or, la clef de la réussite du projet réside bien dans l'implication pleine et entière

Je souhaite que les personnels du RSI soient accueillis le mieux possible et avec la plus grande bienveillance au sein du régime général. Des assurances nous ont été données en ce sens, mais seuls les actes comptent

Des négociations vont avoir lieu entre l'UCANSS et les organisations représentatives du personnel. Il faut qu'elles se tiennent dans un climat apaisé et ne suscitent aucune inquiétude quant à la sécurité juridique de la procédure. Aussi, cet amendement vise à sécuriser la procédure de négociation des accords d'accompagnement entre l'UCANSS et les organisations syndicales des personnels du RSI, en précisant qu'une

Cet amendement rédactionnel déplace une disposition, introduite par nos collègues députés, visant à suspendre, pour les revenus 2018 et 2019 uniquement, la sanction prévue dans le cadre de la procédure de recouvrement des cotisations sur la base d'une déclaration du travailleur indépendant, lorsqu'il existe un écart de plus 30 % entre le revenu déclaré et celui qui est réellement perçu. Ce déplacement permet d'avoir une vision consolidée des initiatives qui seront prises en matière de simplification du prélèvement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

L'alinéa 399 laisse la possibilité aux organismes de recouvrement des cotisations sociales d'opter pour la déclaration mensuelle ou trimestrielle. C'est une simple possibilité, qui relève du bon vouloir de ces organismes. Cet amendement vise à les obliger à proposer aux indépendants d'opter pour un tel dispositif sans limitation de durée afin de préserver leur liberté de choix. Le texte que vous présentez comme ambitieux ne contraindra même pas les organismes de recouvrement à proposer aux indépendants le régime de la déclaration mensuelle ou trimestrielle dès le 1 janvier 2018.

et instaure donc l'autoliquidation comme modalité pérenne de prélèvement des cotisations et contributions sociales. Nous considérons précisément qu'il faut tester cette modalité de recouvrement. Le rapport du Sénat sur le RSI soulignait que ce dispositif ne faisait pas l'unanimité, en particulier auprès des artisans, qui ne souhaitaient pas avoir recours automatiquement à un expert-comptable et redoutaient une augmentation de leurs frais. De leur côté, le RSI et l'ACOSS redoutaient une baisse du rendement du recouvrement et une certaine difficulté pour effectuer des contrôles.

le rapporteur général. Comme le montrent les amendements déposés sur cet article par nos collègues, le véritable enjeu pour les travailleurs indépendants réside bien dans le poids et les modalités de calcul de leurs cotisations sociales. Au-delà du changement de marque- le RSI est incontestablement une marque durablement altérée -, la priorité pour les indépendants est de simplifier le calcul de l'assiette des cotisations et d'améliorer le service de recouvrement. Notre commission a salué l'initiative de lancer une expérimentation sur l'autoliquidation, mais nous considérons qu'elle manque d'ambition. De nombreux rapports ont présenté ces dernières années des propositions visant à simplifier à la fois les modalités de calcul de l'assiette et le service de recouvrement.

Des projets radicalement innovants, comme celui qui a été développé par la start-up d'État « Prélèvement à la source pour les indépendants », ont été proposés. Qu'en pense le Gouvernement ? Est-ce un projet opérationnel ? Et si non, pourquoi ? Les attentes sont grandes, madame la ministre, et je crains que, nourris par la suppression du RSI, de nombreux

de la part du personnel, ce qui est tout à fait légitime. On reprend les mêmes, on recommence, donc soyons attentifs pour faire en sorte que ceux qui ont amené jusqu'à présent une valeur ajoutée peut-être pas suffisamment significative restent quand même dans le dispositif, sinon cela pourrait

une image positive de la transformation. Sinon, pour l'indépendant qui voit les choses de loin, mais qui, bien sûr, participe au dispositif par le biais de ses cotisations,

n'est pas une suppression des régimes unique, donc vous donnez un signal très particulier par rapport à la réforme ambitieuse que vous souhaitez mettre sur pied.

capacité à entendre ces craintes et donc à améliorer le système, tout au long de cette période de transition, période qui garantit aussi, sans doute, la réussite de l'affaire. On voit bien qu'il y a derrière cette transition beaucoup de volonté, notamment par rapport aux salariés du RSI,

la réforme. Combien de fois, les uns et les autres, avons-nous été interpellés sur nos territoires au sujet de situations catastrophiques ? Nous sommes allés au front pour réclamer un regard attentif, empathique, sur les éléments qui nous

aussi au regard des difficultés que pose la transformation, ou en tout cas l'ajustement du RSI au système du droit commun, si je peux m'exprimer ainsi,

nous mettrions en difficulté vis-à-vis des travailleurs indépendants. C'est la raison pour laquelle nous vous faisons confiance et nous disons : allons-y, banco ! Cependant, gardez présentes à l'esprit toutes les interrogations qui ont été formulées ici, ce soir,

amendement de transition entre les articles 11 et 12. Le Gouvernement a annoncé un ensemble de mesures en faveur des travailleurs indépendants, montrant par là une volonté de reconnaissance de ces nouvelles formes d'activité et d'encouragement de la dynamique entrepreneuriale dans notre pays. Certaines de ces mesures trouvent leur traduction législative dans ce PLFSS. Toutefois, la question du risque de requalification du travail indépendant en travail salarié n'est, pour sa part, pas traitée. Il s'agit pourtant d'un risque réel pesant sur les très les très petites entreprises recourant à des travailleurs indépendants, ce qui constitue un frein majeur au développement du travail indépendant et au recours par les entreprises à cette forme de service. Rappelons en effet que les sanctions URSSAF sont particulièrement lourdes en cas de requalification du travail indépendant en travail salarié : les entreprises risquent, comme en cas de travail dissimulé, une remise en cause de l'ensemble des allégements généraux de cotisations sociales sur les cinq dernières années pour l'ensemble de leurs salariés. Or, dans ce domaine, la frontière entre travail salarié et travail indépendant est parfois poreuse. Dans l'attente d'une réponse globale à ce sujet, car je pense qu'il est nécessaire de bien redéfinir clairement les champs des différents termes, il pourrait être proposé que l'URSSAF n'applique pas l'annulation rétroactive sur cinq ans des réductions ou exonérations de cotisations dont l'employeur a bénéficié pour ses propres salariés, sauf, bien entendu, intention frauduleuse manifeste ou récidive, lorsque le redressement concerne la requalification d'une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime. Dans cette période de transition, nous souhaitons que de la souplesse soit introduite, afin de permettre, notamment, que les petites entreprises puissent avoir une vision claire, précise de la définition des différents termes. Tel est l'objet de cet amendement.

d'apporter une réponse à une vraie question. La frontière est effectivement ténue, dans certains cas, entre travail indépendant et travail salarié. Vous souhaitez introduire un aménagement dans l'automaticité de la sanction prévue en cas de requalification d'un travail indépendant en travail salarié. Cette sanction, la suppression du bénéfice de toute exonération de cotisations ou contributions sociales, ne serait pas automatique dans le cas où l'intention de l'entreprise ayant eu recours au travailleur indépendant n'est pas manifestement frauduleuse. Cependant, vous en conviendrez,

Je renvoie d'ailleurs le Gouvernement et nos collègues à la lecture du rapport de la MECSS sur la fraude sociale, rendu l'année dernière, et qui aborde la question de la qualification pénale du travail dissimulé. Pour toutes ces raisons,

toute bonne foi, se voient infliger des sanctions et des modifications du statut du prestataire en salarié, avec toutes les charges sociales qui s'y rattachent.

Je pense qu'il serait plus utile, ou du moins n'est-ce pas incompatible, que l'URSSAF, qui a actuellement une liberté et une marge d'appréciation assez grande, considère les directives de façon beaucoup plus précise, de sorte qu'elle soit amenée à appliquer des règles, et non pas à les interpréter, avec les possibilités qui s'y rattachent. Monsieur Mouiller,

l'esprit de l'amendement est essentiel, et j'espère le retrouver dans le prochain texte. Je retire

Ces mesures renforcent les facilités de paiement octroyées depuis septembre 2017 aux entreprises concernées à la suite d'une instruction ministérielle. L'objectif est d'accompagner sur une période longue, allant jusqu'à décembre 2018, ces entreprises dans leur démarche de redémarrage de leurs activités, et de garantir leur pérennité, vitale pour la vie économique de ces territoires.

C'est bien entendu un vote favorable que j'émettrai, avec le soutien de mes collègues du RDSE, et, je pense, de l'ensemble de

C'est vrai, le monde socioéconomique a toujours tendance à demander plus d'exonérations, etc. Mais pour une fois, dans ce cas précis, c'est justifié, et je voudrais, en mon nom propre,

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est peu dire que le tabac est un véritable fléau en France, puisqu'il totalise à lui tout seul 80 000 décès par an. Si l'on fait la somme des pathologies dues au tabac, que ce soit dans le domaine cardiovasculaire ou dans le domaine du cancer, on s'aperçoit que ce fléau constitue un problème majeur de santé publique. En matière de prévalence, la France détient le triste record d'être le premier pays consommateur de tabac.

cette mesure doit s'accompagner d'un certain nombre d'autres mesures, comme des campagnes de prévention et d'éducation à la santé, tout particulièrement chez les plus jeunes. Il faudra aussi accompagner cette mesure d'un programme de lutte contre la fraude et la contrebande du tabac, faute de quoi la mesure serait bien évidemment inefficace. Je terminerai ce très bref propos en attirant votre attention sur un point particulier : on constate une véritable épidémie, selon le terme employé par une étude récente, de cancers pulmonaires chez la femme. C'est même le seul domaine où l'on peut parler d'épidémie en matière de cancer, tant cette maladie a fortement augmenté chez les femmes. C'est une raison de plus pour s'attaquer à ce fléau au moyen non seulement, c'est l'objet de l'article, de dispositions relatives à la fiscalité, mais aussi, comme le veut d'ailleurs la philosophie générale de ce PLFSS 2018, d'une grande campagne de prévention et d'éducation à la santé.

apporter ma contribution au débat sur cet enjeu important qu'est la lutte contre le tabagisme en abordant une question qui, manifestement, n'a pas du tout été évoquée dans les amendements qui vont venir en nombre tout à l'heure.

du PLFSS correspond globalement aux ambitions du précédent gouvernement, qu'il avait définies dans le programme national de réduction du tabagisme. Je souscris pleinement à cette mesure de santé publique de premier plan. Inutile ici de rappeler le bilan désastreux du tabac : comme le disait notre collègue, 80 000 décès par an, c'est-à-dire à peu près 200 par jour. Je crois qu'il faut aller également au-delà du porte-monnaie et repenser la problématique générale de la consommation en s'intéressant notamment aux incitations culturelles à fumer. Je pense, par exemple, au cinéma, qui valorise la pratique. La Ligue contre le cancer démontre dans une étude que 70 % des nouveaux films français mettent à l'image au moins une fois une personne en train de fumer. Cela participe peu ou prou à banaliser l'usage, si ce n'est à le promouvoir auprès des enfants et des adolescents, qui sont les premiers consommateurs de séries et de films, sur internet notamment. Des solutions doivent être envisagées pour mener une véritable politique de prévention prenant en compte cette sorte de publicité détournée pour la consommation de tabac. J'aurais souhaité, madame la ministre, avoir votre position sur cet état de fait. Je précise, par ailleurs, que cette mesure ne comporte pas de coût financier pour le PLFSS. La

réflexion : je l'ai dit lundi, ce fut l'honneur de Marisol Touraine de mener avec détermination la lutte contre le tabagisme. Toutefois, le très récent Panorama Santé dressé par l'OCDE compte encore 22,4 % de fumeurs en France, contre une moyenne de 18,4 % dans le reste des pays.

pour dissuader de fumer nos concitoyens, notamment les plus jeunes d'entre eux ; nous avons tous en tête les 73 000 décès par an dus au tabagisme. Deuxième réflexion : la France dispose de frontières ouvertes avec des pays qui jouissent d'une fiscalité sur le tabac bien inférieure à la nôtre. Baisse des ventes chez les buralistes ne signifie donc pas baisse de la consommation. Celle-ci s'explique aussi par le déport de l'achat de tabac du circuit officiel vers le marché noir ou, dans les départements frontaliers, vers des achats légaux à l'étranger. Le marché parallèle représente, selon le chiffre des douanes, 27 % du tabac consommé en France. Il serait impératif d'accélérer l'harmonisation fiscale européenne, mais les intérêts des pays sont très divergents. revanche, la traçabilité des cigarettes de l'usine de fabrication jusqu'à la vente au consommateur final doit être mise en place. C'était un objectif du protocole de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, protocole adopté en 2012 à Séoul et élaboré avec le concours de 180 pays. La hausse du prix du tabac doit être assortie d'un plan de lutte contre le marché parallèle, en liaison avec la gendarmerie, la douane, la police et la justice, sans oublier le contrôle des ventes sur internet. Aujourd'hui, en deux clics, me dit-on, il est possible de se faire livrer chez soi des cartouches de cigarettes de l'ancienne marque au paquet rouge. Troisième réflexion réflexion : quelle place, quel rôle éventuel pour la cigarette électronique ? La vapoteuse ne peut-elle pas être envisagée comme un moyen d'arrêt du tabac ? Quatrième réflexion les mesures de prévention mises en place doivent être inventives, notamment en direction des jeunes. Là encore, il faut avoir les chiffres en tête : avec 40 % de fumeurs réguliers chez les 16-25 ans et 19 % chez les adolescents, la France est gravement touchée par ce par ce problème du tabagisme des jeunes. Cinquième et dernière réflexion- monsieur le président, je termine - : quelle diversification, quel avenir pour les 24 000 buralistes en France, dont 43 % sont implantés dans des communes de moins de 3 500 habitants ? Ils constituent

l'on essaye de s'y atteler toujours et encore afin de dissuader au maximum nos concitoyens et nos concitoyennes. Il me semble important de signifier que la fiscalité comportementale doit s'accompagner d'une politique de prévention ambitieuse pour obtenir des résultats en matière de santé publique. Il ne suffit pas, il est vrai, de le décréter. Il y a beaucoup de chemins pour y parvenir, d'autres l'ont dit avant moi.

à augmenter la participation des fournisseurs de tabac au Fonds de lutte contre le tabac, organisme destiné à financer les actions d'information et de prévention du tabagisme.

en termes de prévalence du tabagisme des jeunes, avec un jeune sur trois qui fume quotidiennement et 250 000 adolescents qui entrent chaque année dans le tabagisme.

40 % pour les femmes de 40 ans. On note une explosion- cela a été dit par

Ce que l'on n'a pas dit, c'est le coût sanitaire et le coût social du tabac. Il est évalué par la Cour des comptes en termes de coût social à 120 milliards d'euros par an,

Conscients que les grandes campagnes d'information ne fonctionnent pas, nous devons travailler sur les réseaux sociaux à la dénormalisation de l'image du tabac dans la société, notamment vis-à-vis des jeunes.

qu'augmenter le prix du tabac chez les buralistes, qui ont le monopole de la vente du tabac dans notre pays, sans pour autant lutter très fortement contre la contrebande, voire la contrefaçon, c'est effectivement louper quelque chose vis-à-vis des buralistes auxquels nous devons un accompagnement renforcé. C'est aussi louper quelque chose vis-à-vis d'un trafic qui, en dehors de son aspect très juteux, finance aussi le crime organisé et parfois d'autres réseaux bien plus importants qu'un réseau de cigarettes vendues sous le manteau, si j'ose dire. On l'a vu également pour la contrefaçon, la contrefaçon, parfois les réseaux de contrefaçon peuvent financer des réseaux criminels extrêmement dangereux pour la concorde nationale. Je ne développerai pas davantage ce point. C'est également laisser prospérer des lieux de délinquance dans nos campagnes et nos villes ; chacun peut malheureusement le constater.

d'une transformation qui pourrait être ratée. À ce titre, vous évoquiez, monsieur Daudigny, la cigarette électronique. Il faut avouer que, si l'État n'a parfois pas fait son travail d'accompagnement des buralistes, parfois ce sont quelques-uns des buralistes qui ont refusé les évolutions.

important. Par ailleurs, le nouveau président de la Confédération des buralistes, qui m'a d'ailleurs accompagné toute une journée lors de mon déplacement en Ariège, et que mon administration a déjà rencontré plus de cinq fois depuis son élection le mois dernier, travaille activement dans un esprit de grande responsabilité. Il n'est pas du tout dans l'idée du Gouvernement de nier cette activité professionnelle très importante et que l'on doit désormais aider à se transformer. somme, monsieur le sénateur, je crois que le Gouvernement a pris en considération les demandes des parlementaires, notamment en ce qui concerne la lutte, très importante, contre la contrebande et la contrefaçon.

Si nous ne sommes pas opposés par principe à une hausse, il conviendrait pour autant de ne pas faire de la hausse du tabac un élément que l'on retrouve chaque année dans le projet Deux éléments nous conduisent à proposer la suppression de l'article 12. Tout d'abord, comme la corrélation entre la hausse des prix du tabac et la baisse du nombre de fumeurs n'est pas établie, pourquoi renouveler sans cesse une mesure qui n'a pas prouvé son efficacité ? Ensuite, les hausses successives de ces dernières années ont eu pour conséquence de favoriser l'achat de produits du tabac dans les pays limitrophes, en particulier en Andorre, et d'encourager le marché parallèle. Nous appelons le Gouvernement à instaurer un moratoire sur les prix du tabac et à diversifier les pistes permettant de lutter contre la consommation excessive de tabac.

cette fin de séance. Mais la patience est mère de toutes les vertus : ce sera pour demain ! Les buralistes ont une part active dans le maillage du territoire dans le commerce de proximité. Sur les 24 000 buralistes en France, qui emploient quelque 100 000 personnes, 43 % exercent dans des communes de moins de 3 500 habitants. Il s'agit donc d'une activité essentielle à la vie de nos régions et de nos départements. Une hausse du prix du tabac fragilise encore un peu plus l'équilibre précaire de nos territoires, notamment dans nos régions frontalières. des buralistes est déjà gravement menacée par une forte contrebande qui compromet les actions entreprises pour la protection de la santé des Français. Nous savons bien qu'une hausse du prix du tabac profite grandement à cette contrebande que vos frontières passoires, désormais inexistantes, ne sont malheureusement pas en état d'endiguer. Contrebande et contrefaçon- vous l'avez évoqué vous-même, monsieur le ministre -créent et développent une insécurité sanitaire. Ainsi, votre politique se fait au détriment des buralistes et n'a qu'un effet limité sur la consommation de tabac des Français. En effet, l'expérience ne démontre pas

de paquets de cigarettes de contrebande et de contrefaçon. Je peux vous assurer sans exagération aucune qu'à Marseille, sur la Canebière, qui devrait être un véritable sanctuaire, la vente de paquets de cigarettes de contrebande et de contrefaçon se fait non pas sous le manteau, mais à la vue et au su de tous, et ce à moins de 100 mètres du commissariat central, malgré l'investissement des policiers. Eh bien, ce trafic en plein jour ne cesse toujours pas De plus, une fois encore, la hausse du prix du tabac est une mesure fiscale qui va pénaliser les Français et, notamment, les plus modestes d'entre eux. Il est possible d'avoir une politique préventive sans matraquer fiscalement les fumeurs. La Suède, par exemple, a obtenu de bons résultats. Axons donc nos efforts sur la prévention et la pédagogie, en particulier auprès des plus jeunes, et évitons d'étrangler fiscalement les fumeurs et de mettre en péril une profession qui participe activement au lien social de nos territoires